au règlement. Sur le fondement de l'article 36 de notre règlement, le groupe communiste républicain citoyen et écologiste souhaite interpeller le président du Sénat et le ministre chargé des relations avec le Parlement sur le respect du droit d'amendement des groupes parlementaires. Le 18 octobre dernier, le Président de la République a déclaré qu'une réforme constitutionnelle s'imposait sur le droit d'amendement, car nous aurions « tous collectivement contribué à une inflation législative » et à « l'illisibilité de notre droit ».

J'appelle solennellement les groupes politiques à prendre conscience de la réduction du droit d'opposition et du droit constitutionnel d'amendement, sachant que notre temps de parole pour défendre les amendements a été parallèlement diminué. Nous avons la désagréable impression que le but est d'en finir au plus vite avec l'examen de ce PLFSS. Les sommes impliquées sont pourtant bien plus importantes que dans le cadre du PLF, pour lequel un examen de trois semaines

sur l'article. L'article 4 prévoit un allégement de la taxe sur la vente en gros des spécialités pharmaceutiques. Si les grossistes-répartiteurs ont été en première ligne pour la fourniture des masques et des vaccins à nos concitoyens, le Gouvernement le Gouvernement propose un allégement de 5 millions d'euros pour les laboratoires pharmaceutiques et de 30 millions pour les grossistes-répartiteurs. Cela représente 35 millions de recettes fiscales en moins pour la sécurité sociale. On peut s'interroger sur les contreparties demandées par l'État. Selon l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, 2 400 médicaments auraient manqué en 2020, soit quatre fois plus qu'en 2016. Notre groupe avait déposé un amendement, malheureusement déclaré irrecevable, tendant à faire passer de deux à quatre mois l'obligation de stock des laboratoires et des grossistes-répartiteurs. Nous souhaiterions savoir si des mesures de lutte contre les pénuries de médicaments et de produits de santé leur sont imposées en contrepartie.

Cela pose une véritable question de choix économiques, voire de choix éthiques. Le Gouvernement préfère accorder une baisse de fiscalité à des groupes pharmaceutiques incapables de produire un vaccin contre le covid-19

dont l'objectif est de restaurer de manière mineure leur marge de 0,25 point. Deuxièmement, cette baisse des recettes est estimée, pour la sécurité sociale, à 35 millions d'euros en 2021, puis à 37 millions d'euros en 2022 ; elle n'est pas compensée pour l'assurance maladie.

L'allégement de la taxe sur la vente en gros de médicaments est l'une des trois mesures envisagées par le Gouvernement pour restaurer les marges des grossistes-répartiteurs. Les deux autres consistent en l'augmentation par arrêté des marges réglementées et en l'instauration d'un forfait spécifique pour la distribution de médicaments conservés au froid. Par ailleurs, cet allégement bénéficiera très majoritairement aux grossistes-répartiteurs, pour 85 %. Les laboratoires qui réalisent des ventes directes aux officines restent encore très minoritaires dans le circuit de distribution en ville.

qui assurent la répartition, distribuant une large gamme de médicaments, des, lesquels concentrent leur activité sur la vente directe de quelques références pourvoyeuses de marges importantes et n'assurent pas les missions de service public. Attirés par la rentabilité du marché du médicament, les ont, la plupart du temps, une activité d'import-export sur des produits contingentés par les laboratoires. Dès lors, ils ne respectent ni l'obligation de disposer d'un stock de médicaments

monsieur le ministre,

Compte tenu des économies réalisées par les organismes complémentaires pendant la crise et, dans le même temps, de l'augmentation inédite des dépenses de la branche maladie, il nous paraît naturel de porter cette contribution à 1 milliard d'euros, au lieu de 500 millions. Nous demandons aux mutuelles de consentir un effort supplémentaire exceptionnel, une action de solidarité dans un contexte tout aussi exceptionnel où les comptes de la sécurité sociale sont entraînés Quel est l'avis de la commission ?

Considérant que les économies de constatation dues à différents facteurs liés à la crise du covid rendaient légitime la contribution des organismes complémentaires au financement de la sécurité sociale, Oliver Véran et moi-même avions demandé

Force est de constater que tel n'est pas le cas puisque la quasi-totalité des organismes complémentaires a annoncé une augmentation de leurs tarifs, à des niveaux qui semblent même supérieurs à l'inflation.

sur les organismes complémentaires d'assurance maladie à 1 milliard d'euros, au lieu des 500 millions d'euros prévus l'an dernier par le PLFSS. L'an dernier, cette mise à contribution exceptionnelle des organismes complémentaires d'assurance maladie au profit de la branche maladie s'expliquait par le niveau des économies réalisées durant la pandémie, à hauteur d'environ 2 milliards d'euros. Depuis, la situation a évolué, et le Gouvernement a accepté de diviser par deux la contribution des complémentaires pour tenir compte de l'augmentation des dépenses de santé, en contrepartie d'une modération des tarifs. L'annonce par certains organismes d'une hausse de leurs tarifs au niveau de l'inflation a remis en cause l'engagement pris par les organismes complémentaires de maintenir leurs tarifs au même niveau que l'an dernier, en échange de la réduction de la taxation. Nous tirons trois conclusions de cet épisode. Tout d'abord, il est difficile de négocier avec les organismes complémentaires,

tarifs, et fait peser sur les adhérents les coûts supplémentaires, ce qui est complètement injuste. Enfin, cette taxe symbolique pose avant tout la question du financement de la sécurité sociale. Nous gardons à cet égard un un intérêt certain pour une « grande sécurité sociale », à condition que celle-ci repose sur les cotisations des salariés et des employeurs et assure un remboursement à 100 % des dépenses de santé. La

126. Cet amendement a pour objet de fixer une compensation à son coût réel du budget réel de l'Agence nationale de santé publique (ANSP), plus connue sous le nom de Santé publique France.

pour répondre à la crise sanitaire- masques, tests, etc. En 2021, une nouvelle augmentation de 4,3 milliards d'euros a abondé le budget de l'Agence. Cela confirme la pertinence de l'analyse du Sénat, qui s'était opposé au transfert de l'ANSP à la sécurité sociale au motif que cette agence remplit des missions de l'État. En outre, le Gouvernement a profité de ce transfert pour s'exonérer de toute demande d'autorisation du Parlement quand il a augmenté massivement les crédits de l'Agence par de simples arrêtés ministériels. Il convient que la sécurité sociale soit compensée à due concurrence des coûts extraordinaires intervenus dès la première année du transfert. Par la suite, la question du recalibrage de cette compensation se posera. Je reprends à mon compte l'argumentation de notre rapporteure. La situation nous apparaît aujourd'hui inacceptable. Nous considérions au moment où a été décidé le transfert de Santé publique France du budget de l'État vers celui de la sécurité sociale qu'il s'agissait d'une erreur, puisque cette agence, qui remplit des missions de l'État, devait demeurer à ce titre dans le budget de l'État. La crise sanitaire nous a malheureusement donné raison : ce transfert a considérablement plombé les comptes de la sécurité sociale, puisque le budget de Santé publique France a augmenté de plus de 4 milliards d'euros. Plutôt que d'accepter

de la santé. Ce débat, que nous avons eu les années précédentes, met au jour des désaccords récurrents entre le Sénat et le Gouvernement. Nous considérons qu'il est logique que le budget de Santé publique France, même s'il est plus important du fait d'une épidémie, relève de la sécurité sociale.

les comptes de la sécurité sociale puissent être équilibrés au prix d'un déséquilibre durable des comptes de l'État. De la même manière, je ne crois pas que les comptes de l'État puissent être équilibrés au prix d'un déséquilibre durable des comptes de la sécurité sociale. Le contribuable et l'assuré social sont

D'une part, derrière cette annonce, le Gouvernement a transféré la dette à la Cades, en laissant à la sécurité sociale le soin de rembourser une dette qui n'était pas la sienne puisqu'il s'agissait en majorité de dette immobilière.

doit amortir une dette sociale. L'investissement et l'amélioration des conditions de fonctionnement et d'exercice des hôpitaux relèvent d'une logique de protection sociale. Il est donc tout à fait logique et cohérent que les modalités de financement soient celles que nous avons prévues. Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements identiques.

outre, nous considérons que la perte d'autonomie des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées est liée à l'état de santé, et que les dépenses doivent donc relever de l'assurance maladie.

un grand service public national de la perte d'autonomie et de l'accompagnement, avec l'ensemble des structures d'aide à domicile et du secteur médico-social. Or le Gouvernement refuse de faire payer les dépenses liées à la perte d'autonomie aux entreprises et aux revenus financiers, qui accumulent des richesses sur le dos de nos aînés, ce que nous désapprouvons. D'où cet amendement de suppression

à tirer les conséquences de plusieurs données ou décisions relatives aux prévisions de recettes, aux objectifs de dépenses et au tableau d'équilibre par branche du régime général et des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale pour 2021.

à une interpellation de M. Mouiller - ; et à tenir compte d'une révision à la hausse de la dynamique des dépenses de soins de ville, à hauteur de 500 millions d'euros par rapport au montant inscrit dans le texte initial.

Nous ne nous opposons pas aux dépenses rendues nécessaires par la crise sanitaire, cela va de soi, mais justement, parce que nous agissons en responsabilité, nous ne pouvons nous borner à constater les dépenses. Il s'agit d'une question de respect des droits et des missions du Parlement.

Vous vous en souvenez sans doute, mes chers collègues, le PLFSS pour 2020 prévoyait déjà l'unification des retraites complémentaires d'une partie des régimes spéciaux spéciaux et des employeurs publics. Selon l'étude d'impact de ce projet de loi, ces « différentes étapes permettr[aie]nt que l'unification du recouvrement des cotisations sociales constitue utilement un acquis pour la mise en oeuvre future de la réforme des retraites ».

amendement tend à prévoir que les accords conclus pour préciser les modalités, conditions et garanties applicables à ces salariés dans le cadre de leur transfert s'appliqueront jusqu'au 31 décembre 2025.

En raison de la crise sanitaire, plus d'un million de nos concitoyens ont basculé dans la pauvreté. Absolument ! Toutes les associations de soutien aux personnes en difficulté font d'ailleurs état d'une explosion de la demande d'aide alimentaire ou d'accompagnement social, et les démarches d'accès à la couverture maladie Or, en raison du processus de dématérialisation engagé depuis plusieurs années et des conditions sanitaires, de nombreuses personnes ne maîtrisant pas toujours les outils numériques se trouvent aujourd'hui dans l'impossibilité d'obtenir des réponses à leurs questions ou de l'aide dans leurs démarches.

avec un versement anticipé, vous préservez, certes, le budget des familles, mais vous prenez le risque d'une augmentation du nombre d'erreurs, de rectifications ou de trop-perçus. En effet, en 2022, les familles bénéficieront d'exonérations de cotisations sociales calculées sur les aides versées et déclarées en 2021.

Cette mesure permettra de limiter l'avance de trésorerie qui peut parfois représenter, pour nombre de citoyens, un obstacle à l'utilisation de services pourtant essentiels. Simplifier les outils existants dans le domaine des services à domicile

mesure. L'amendement n° 129 tend ainsi à préciser que le dispositif CESU tiers payant ne concerne que les particuliers employeurs et les particuliers recourant à un mandataire, à l'exclusion des particuliers clients de prestataires. Le CESU tiers payant permet aux conseils départementaux de prendre en charge les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi d'un salarié à domicile par un allocataire de l'APA à domicile ou de la PCH sous forme de titre préfinancé, au lieu de lui verser ces aides par virement postérieur au paiement du salaire. L'amendement n° 130 a pour objet de préciser que le nouveau dispositif de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne, créé à l'article 11

Cet amendement vise à permettre à tous les foyers ayant recours à des services à la personne de bénéficier de cette mesure dès le 1 janvier 2022. Il s'agirait d'autoriser les structures de services à la personne à mettre en place un processus transitoire leur permettant d'offrir, dès le 1 janvier 2022, un équivalent du crédit d'impôt instantané à leurs clients. Pour ce faire, elles consentiraient, sur les trois premiers mois de l'année 2022, à faire l'avance de trésorerie du crédit d'impôt

? J'entends bien votre préoccupation, mon cher collègue, mais seule l'avance du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile sera généralisée aux particuliers recourant à un mandataire ou à un prestataire au 1 avril 2022, tandis que les aides sociales ne leur seront avancées qu'à partir de 2023. Aussi n'est-il pas envisageable de rembourser les sommes prises en charge au titre de ces dernières dès le 1 avril 2022. Avis défavorable.

dispositif fiscal et de celui des cotisations sociales auxquelles sont assujetties les associations à but non lucratif.

mesure où il s'agit d'un petit problème essentiellement administratif de déclaration, avec un enjeu financier sans doute très faible pour la sécurité sociale, le Gouvernement pourrait peut-être nous éclairer sur ce qu'il conviendrait d'entreprendre pour faciliter la vie des organismes et associations concernés. Quel

des non-résidents d'un État tiers à l'Europe constitue une réelle discrimination face à l'impôt et décourage l'investissement en France de nos compatriotes installés à l'étranger.

à adhésion volontaire, comme la Caisse des Français de l'étranger (CFE), soit au système de protection sociale de leur pays de résidence. Cette situation les conduit donc à subir une double imposition

Au nom du principe d'équité fiscale, l'exonération de CSG et de CRDS devrait être généralisée à tous les non-résidents, où qu'ils habitent.

revenus en France ? Cela n'a aucun sens. En termes d'équité fiscale, c'est totalement indéfendable. Or c'est bien ce dont il s'agit ici : les uns paient la GSG-CRDS ; les autres pas.

mais aussi aux étrangers installés en France. Tel doit particulièrement être le cas de la CSG et de la CRDS sur les revenus patrimoniaux, qui permettent de faire participer le capital au financement de la solidarité. De ce point de vue, la cohérence de certains signataires d'amendements prête d'ailleurs à interrogation. européenne (CJUE) contraint la France à exonérer les personnes relevant d'un autre régime de sécurité sociale européen. Mais un autre arrêt de la même Cour souligne expressément qu'il est loisible à la France de faire participer à la solidarité nationale les autres personnes non inscrites à sa sécurité sociale. La commission préfère donc s'en tenir aux obligations juridiques de la France, sans aller plus loin.

hausse exceptionnelle, pour l'année 2022, de la taxation des revenus du capital- produits de placement et patrimoine -pour répondre aux besoins de financement de la crise sanitaire. Alors que la CSG des revenus d'activité et de remplacement- salaires et pensions de retraite -a augmenté de 1,7 en 2018 pour financer la baisse de cotisations sociales chômage et maladie, le taux applicable aux revenus du capital- produits de placement et patrimoine -n'a augmenté que de 1 point. proposent donc d'augmenter la CSG sur les revenus du capital de 1,4 point. Une telle progression permettrait un rendement supplémentaire de 1,5 milliard d'euros au profit des organismes de sécurité sociale. Ces sommes pourraient être exceptionnellement affectées à la gestion de la crise sanitaire

et les agents publics. Après la crise sociale de 2019, le Gouvernement a fixé un seuil de 2 000 euros mensuels en deçà duquel les retraités ne sont pas assujettis au taux de CSG revalorisé- 6,6 % au lieu de 8,3 %. Nous proposons de retenir un seuil de 3 000 euros mensuels, ce qui permettrait de redonner du pouvoir d'achat aux retraités, qui en ont besoin en ce moment. Quel

il n'est pas d'interdit d'observer que ce sont les revenus des actifs, et non ceux des retraités, qui ont subi les conséquences de la récente crise. Il est donc difficile d'augmenter l'écart, à revenu égal, entre la CSG acquittée par les actifs et celle acquittée par les retraités, ainsi que le proposent

Cet amendement tend à créer un abattement fiscal au profit des retraités agricoles qui décident de mettre en location une partie ou l'intégralité de leurs exploitations- opération plus communément appelée « fermage

Aussi, le fermage est devenu une option pour les agriculteurs retraités qui cherchent à obtenir un complément à la faible pension de retraite qu'ils perçoivent. Toutefois, cette option se heurte à un niveau d'imposition très important

qui conduit à une tentation de plus en plus grande d'artificialiser ces terres, dans l'optique de vendre au prix des terrains à bâtir. Or, pour un grand nombre de retraités agricoles à la pension très modeste, ces terres ont représenté, pendant leur période d'activité, leur outil de travail,

sur ceux appliqués aux retraités, ce qui permettrait de reconnaître la véritable nature de ces revenus, à savoir celle d'un complément de retraite et non d'un investissement à caractère patrimonial.

dont l'assiette, à la différence de l'impôt sur le revenu, n'est encore pas trop entamée par les niches sociales. Il importe de préserver cet état de fait pour conserver l'intelligibilité et l'efficacité de cet impôt. En outre, l'instrument le plus à même de soutenir les revenus des retraités agricoles n'est pas un abattement de CSG, qui entamerait l'équilibre déjà très fragile des comptes de la sécurité sociale, mais une hausse des petites pensions.

1 % assise sur les revenus des capitaux mobiliers, pour financer la cinquième branche. En effet, la création de cette branche n'a pas donné lieu à un financement pérenne. Le rapport Libault

Le prélèvement envisagé est très modéré, puisqu'il est bien inférieur aux économies que les grandes fortunes ont réalisées dans le cadre de la en 2017.

rapports présentent d'autres sources de financement. Cet amendement vise à reprendre l'une des propositions du rapport Vachey pour financer l'autonomie, à savoir la mise en place d'une contribution assise sur les droits de succession et de donation les plus importants, c'est-à-dire lorsque

créer cette nouvelle source de recettes.

Sur ces amendements

Face à l'urgence sanitaire et à la nécessité de trouver de nouvelles recettes pour financer notre système de santé, nous proposons de mettre à contribution les montants versés aux actionnaires aux taux actuels des cotisations sociales employeurs de la sécurité sociale.

Cet amendement de repli vise donc à créer une contribution de 2 % sur les dividendes versés aux actionnaires. Il nous paraît juste de mettre à contribution les actionnaires plutôt que les salariés et les retraités,

participent à l'adaptation de la société au vieillissement. L'objectif est d'augmenter le budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie afin de mieux prendre en charge les situations de perte d'autonomie, tout en garantissant une égalité de traitement sur le territoire national. Je rappelle que les dividendes ne sont que rarement réinvestis en France : ils enrichissent des fonds de pension, des gestionnaires d'actifs et des fonds vautours. Ces dividendes sont symptomatiques d'un modèle qui repose sur la création de valeur actionnariale à court terme et néglige bien trop souvent toute responsabilité sociale, pour ne rien dire des responsabilités environnementales. Les grandes entreprises et leurs actionnaires doivent participer à l'effort commun de solidarité et

favorable sur cet amendement,

Le scrutin est clos.

et d'activité physique adaptée par les complémentaires santé doit être encouragé- nous sommes unanimes sur ce point -, il convient de rappeler que la taxe de solidarité additionnelle finance la complémentaire santé solidaire et que les dépenses des complémentaires santé santé ont été réduites par la crise sanitaire. Il ne semble donc pas judicieux de prévoir des allégements de TSA à l'heure où les complémentaires santé vont prendre toute leur place dans le redressement des comptes de la sécurité sociale. Avis

permettant la prise en charge de l'activité physique adaptée.

réservant ainsi le régime social et fiscal afférent aux seuls agents dont les employeurs auront fait le choix de cet unique dispositif de couverture. Là où l'ordonnance visait à réduire les inégalités entre agents publics et salariés du secteur privé,

nous est soumis comporte une ambiguïté, qu'il convient de lever. Il est ainsi proposé d'indiquer de façon explicite que le dispositif d'exonération prévu est bien lié à la participation obligatoire de l'employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents, et non à un seul type de contrat.

%. La participation obligatoire à 50 % ne s'appliquera qu'à compter de 2024 pour les agents de la fonction publique d'État et de 2026 pour les agents hospitaliers et territoriaux.

En outre, les contrats collectifs obligatoires sont objectivement les plus solidaires. Si l'adhésion n'est que facultative, en effet, les plus jeunes et les mieux portants, dont le risque est minoré et qui font baisser la prime de tout le monde, ne souscriront pas. Dès lors, je soutiens l'équilibre qui a été trouvé dans l'ordonnance. J'en rappelle le dispositif : d'une part, tous les agents publics adhérant à une complémentaire bénéficient d'une participation de leur employeur, étant entendu que tout le monde est avantagé dans le nouveau système par rapport à la situation antérieure

et que nous avons mis en place cette trajectoire progressive en accord avec les représentants des employeurs de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

lent, je suis d'accord avec Mme la rapporteure sur un point : il faut que les contrats soient obligatoires et collectifs. C'est essentiel

agi de mettre en place ce nouveau droit et cette convergence avec le secteur privé, favorable aux agents publics, il a été dit et démontré par lesdits employeurs que le caractère soutenable de la montée en puissance nécessitait ces deux ans.

n° 45 rectifié. L'harmonisation du régime fiscal et social des contributions des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des agents et la création d'un mécanisme d'exonération fiscale et sociale en la matière rendent est, d'adapter le dispositif et d'encourager la couverture la plus large des agents de la fonction publique, indépendamment du type de contrat de PSC retenu par l'employeur public.

L'objet de cet amendement est de garantir un maintien de la rémunération pour les personnes qui assumeraient la charge d'un proche en perte d'autonomie. Ce dispositif s'imposerait aux conventions et aux accords collectifs, comme le prévoit l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

le rehausser à hauteur du SMIC, garantissant ainsi la pleine effectivité de ce nouveau droit en consolidant le niveau de son indemnisation. La situation des personnes en congé de proche aidant va donc connaître une amélioration significative et le recours à cette prestation Il nous paraît par ailleurs prématuré d'envisager une prise en charge de la perte de revenu non couverte par l'AJPA ou par l'AJPP puisque l'impact d'une telle réforme sur le secteur de la protection sociale complémentaire ne peut pas être connu pour

Cet amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subies. permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins. Ce n'est pas sans conséquence pour les assurés, qui voient leur reste à charge varier en fonction du professionnel auquel ils s'adressent. C'est pourquoi il est proposé, au travers de cet amendement, de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé par une limitation du niveau possible de différenciation des remboursements.

est l'avis de la commission ? Cet amendement vise à revenir à la logique initiale du contrat solidaire et responsable en mettant surtout fin aux avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les organismes complémentaires sur la taxe de solidarité additionnelle.

est 27 % plus élevé qu'en Allemagne, 37 % plus élevé qu'en Italie et 75 % plus élevé qu'en Pologne. Les fruits et légumes, majoritairement importés en France, proviennent de pays qui n'ont pas les mêmes règles et les mêmes contraintes environnementales que nous.

Quel est l'avis de la commission ?

un agriculteur sur deux y est adhérent. Ces coopératives ont permis de promouvoir diverses formes de mutualisations et ont été pionnières pour le développement des groupements d'employeurs dans la coopération agricole. Cependant, elles sont toujours exclues du bénéfice de l'exonération visée à l'article L. 741-16 du code rural

serait sans doute une erreur

l'interdiction de délocaliser des activités à l'étranger si cela entraîne une diminution du nombre d'emplois en France ; et la remise d'un rapport annuel faisant état de la trajectoire de la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon de 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national.

patronales pour l'assurance maladie à des critères sociaux et écologiques afin d'engager toutes les forces productives dans une transition sociale et écologique, vers une société plus juste et vivable pour les générations futures. Houerou. Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise également à conditionner les allégements de cotisation patronale à des obligations en matière sociale, environnementale et fiscale pour les entreprises dont la taille correspond ou excède le seuil européen de l'entreprise moyenne. Ces obligations sont les suivantes : premièrement, la remise d'un rapport annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon de 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre deuxièmement, l'obligation de ne pas délocaliser des activités à l'étranger entraînant une diminution des emplois en France ; troisièmement, la mise en place d'une égalité salariale entre les femmes et les hommes. Le non-respect d'au moins l'une de ces trois obligations entraînerait un remboursement du bénéfice de l'allégement de cotisation patronale et le paiement d'une sanction pécuniaire définie par décret. Quel

un avis défavorable. Quel est l'avis du Gouvernement ? Le débat sur la conditionnalité des aides sociales, comme des aides fiscales, d'ailleurs, a eu lieu à plusieurs reprises à l'occasion de chacun des textes financiers. J'ai donc déjà eu l'occasion de dire pourquoi le Gouvernement était favorable à des dispositifs sans conditionnalité excessive. Concernant les allégements de charges en particulier, le Gouvernement, lorsqu'il a transformé ce crédit d'impôt en allégement général, s'est inspiré du dispositif qui préexistait depuis 2013, c'est-à-dire l'absence de conditionnalité. J'émets

Cathy Apourceau-Poly. Mon collègue Pascal Savoldelli a proposé, dans notre amendement précédent, de fixer des contreparties à la suppression des cotisations sociales à la branche famille. C'était en quelque sorte notre amendement de repli puisque celui-ci vise à rétablir complètement les cotisations des entreprises à la branche famille de la sécurité sociale. Ce manque à gagner, évalué à 20 milliards d'euros, remet en cause le principe même des cotisations des entreprises à la sécurité sociale. Surtout, cette suppression des cotisations patronales en deçà du SMIC remet en question le fondement idéologique de notre système de protection sociale, qui consiste à partager la valeur créée au sein de l'entreprise. Les cotisations sociales sont la part socialisée du salaire. La suppression des cotisations patronales revient sur le principe du paritarisme de financement de la sécurité sociale. En rétablissant ces cotisations à la branche famille, la sécurité sociale pourrait ainsi envisager l'indemnisation à 100 % au niveau des salaires des congés de maternité de paternité, ou la création de 100 000 places en crèche supplémentaires. Voilà des exemples d'une utilisation plus efficace et pertinente de ces 20 milliards d'euros ! Quel

estimations. Cet amendement pose néanmoins une vraie question sur l'efficacité d'un allégement de cotisations allant aussi loin dans l'échelle des salaires. Le Gouvernement pourrait sans doute engager une réflexion utile sur le reformatage des allégements, éventuellement à produit constant.

est inefficace en termes de créations d'emplois et de compétitivité. Il est également coûteux pour les finances sociales, avec une perte de recettes de 8 milliards d'euros pour la branche famille. Je pense, madame la rapporteure générale, que vous êtes sensible à ce manque à gagner. Les auteurs de

que constitue la prévention plus efficace de l'apparition des souffrances liées au travail. Nous proposons, au travers de cet amendement, de meilleures évaluation et prévention du burn-out grâce à un mécanisme de malus pour les employeurs n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer le risque avéré d'épuisement professionnel. Nous proposons également de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises, qui présente une sinistralité anormalement élevée. je partage la volonté des auteurs de l'amendement de diminuer les risques professionnels dans l'entreprise, je rappelle que les cotisations que versent les employeurs pour financer la branche AT-MP

La part variable du taux de cotisation AT-MP atteint presque 70 % en moyenne. Plutôt que de pénaliser les employeurs, qui remplissent déjà un document unique d'évaluation des risques professionnels substantiel, il importerait de mieux les accompagner en matière de prévention, comme l'a rappelé Pascale Gruny dans son rapport. C'est en ce sens qu'a été adoptée la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, qui a notamment transformé les services de santé au travail en services de prévention et de santé au travail. Enfin, les entreprises supportent un poids manifestement excessif en matière de cotisations AT-MP : les excédents cumulés devraient dépasser les 5 milliards d'euros fin 2022. elles supportent déjà une série de majorations, dont celle destinée à financer le transfert à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des AT-MP. Pour toutes ces raisons, l'avis est défavorable.

services font preuve d'un fort engagement d'adaptation et d'abnégation durant la crise sanitaire que nous traversons. Ces structures d'aide employant des salariés qui interviennent au domicile des personnes fragiles peuvent bénéficier d'une exonération des cotisations patronales, à condition d'être gérées par des centres communaux (CCAS) ou intercommunaux d'action sociale public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat de communes, ils en sont exclus. Cela conduit à une situation injuste et inégalitaire. Ces structures doivent acquitter des charges supplémentaires, alors même que leur équilibre budgétaire est fragile et qu'elles assurent au quotidien les mêmes missions au service d'un même public avec des agents au même statut. L'objet de cet amendement est de donner de la cohérence entre les différents modes de gestion, et donc de rendre éligibles aux exonérations de charges patronales les agents travaillant pour des services d'aide à domicile gérés par des communes ou par des EPCI. Quel est l'avis de la commission ?

Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale bénéficient de l'exonération d'aide à domicile pour ne pas désavantager les agents de ces organismes par rapport aux autres secteurs, notamment au secteur privé. Le champ d'application a été validé par le Conseil constitutionnel une décision le 5 août 2011. Dans sa décision, le Conseil a considéré que le législateur entendait ainsi favoriser la coopération intercommunale spécialisée en matière d'aide sociale. Je ne conteste évidemment pas que les agents des EPCI peuvent remplir les mêmes tâches d'aide à domicile que ceux des CCAS et des CIAS. Il n'en reste pas moins que les EPCI

Pour nous, le rôle de l'État est tout autre : ce dernier doit garantir la juste participation de toutes et tous à l'élaboration d'un projet collectif qui profite à l'ensemble de la société, ce qui implique de garantir un service public permettant à chacun de jouir de ses droits fondamentaux, en l'occurrence le droit à un égal accès aux soins. Si nous ne luttons pas contre ce manque à gagner, nous ne serons pas en mesure de renforcer la résilience de notre système de santé face aux prochaines pandémies et de préparer l'ensemble du système de soins à affronter le vieillissement de la population. Nous demandons la fin de la transposition du CICE dans le droit, parce que ce dispositif s'est montré inopérant socialement et parce qu'il faut rendre à l'État les moyens de maintenir nos structures de soins et de garantir l'investissement dans la santé.

Nous estimons que les dispositifs d'exonération de cotisations sociales favorisent les contrats courts imposés aux femmes. Pour y remédier, il nous faut être un peu plus fermes. Nous proposons, dans une logique de contrepartie, de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales dans les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en

en Bretagne, avec à la fois du personnel mis à disposition par les conseils départementaux pour exercer des missions traditionnellement d'intérêt général et de plus en plus de salariés sous contrat de droit privé.

est l'avis de la commission ?